madame la présidente.

d'un travail plus global sur les différents instruments de gestion de futures urgences sanitaires. Nous souhaitons donc le maintien de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa forme actuelle.

; je vais donc développer celle-ci. Vous voulez supprimer l'article 4 ; il a pourtant été écrit pour vous et vos semblables, les ministres effet, si on laisse l'article L. 3131-1 du code de la santé publique en l'état, vous ne pourrez jamais rien en faire. Or nous espérons tous que vous n'aurez pas à revenir devant le Parlement pour un nouvel état d'urgence sanitaire. Le 31 décembre 2021, le régime

totalement inopérant, mal rédigé, et qui donnerait, si l'on en faisait une interprétation extensive, des pouvoirs exorbitants au ministre de la santé, que même le Premier ministre ne pourrait pas exercer sans une habilitation législative- la preuve : le Gouvernement nous a demandé, par la loi 23 mars 2020, d'établir un régime de l'état d'urgence pour fonder l'exercice de pouvoirs exceptionnels en cas de pandémie. Monsieur le secrétaire d'État, pensez que vous pourriez un jour avoir besoin d'un article L. 3131-1 du code de la santé publique qui soit

La protection des données est un enjeu fondamental, particulièrement lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel ou de données de santé. L'encadrement que nous avions introduit allait jusqu'à prévoir la suppression de ces données dans des délais courts, toujours de quelques mois après l'issue de la crise sanitaire.

ans. Je tiens à rassurer sur ce transfert et à souligner sa pertinence. Le SNDS est un système sûr et le dispositif que j'ai proposé, que la commission des lois a retenu- je remercie M. le rapporteur d'avoir accepté les amendements que j'ai présentés au nom de la commission des affaires sociales

de recherche. J'insiste ici sur la pertinence de ces transferts. Les données recueillies durant la pandémie représentent un fort potentiel pour la recherche médicale, notamment en matière de modélisation de la diffusion épidémique, et donc aussi pour l'évaluation de nos politiques de santé publique. Il ne faut pas avoir peur de l'exploitation des données de santé : je crois en l'utilité des données recueillies durant la pandémie de covid-19 pour mieux nous préparer à de futures épidémies. L'amendement

des données personnelles liées à la pandémie de covid-19, position que le ministre de la santé avait soutenue le 20 janvier dernier devant les députés.

Si la recherche sur le virus est indispensable, elle ne doit pas remettre en cause l'anonymat de ces données. Or, en croisant les données des différents systèmes d'information, il est possible de retrouver l'identité des personnes auxquelles elles appartiennent. Je rappelle que les hôpitaux français ont été particulièrement touchés par les cyberattaques et que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information travaille actuellement à des obligations de sécurité plus rigoureuses afin de protéger les données de santé de nos concitoyens. Les garanties ajoutées par la commission des lois du Sénat, qui limitent l'accès à ces données et leur traitement aux services de l'État et des établissements publics, sont positives mais insuffisantes pour nous rassurer Tout cela présente un réel danger pour les libertés individuelles et pour la nécessaire confidentialité des données de santé. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l'article 5. Quel

Nous y avons ajouté un amendement qui nous a été inspiré par les règles appliquées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont l'objet est de prévoir un droit d'opposition

votre amendement vise à empêcher le rassemblement des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information destinés à la lutte contre l'épidémie de covid-19 au sein du système national des données de santé. Le SNDS rassemble et met à disposition les données issues des systèmes d'information mis en oeuvre dans le secteur de la santé afin de contribuer notamment- vous avez évoqué ce point -à la recherche,

de meilleure compréhension de l'épidémie et de ses impacts sur le système de santé, il nous apparaît nécessaire de prévoir expressément que les données ainsi collectées seront rassemblées au sein du SNDS et seront soumises aux dispositions du code de la santé publique qui encadrent celui-ci. Sans cette disposition,

elles garantissent un haut niveau de protection. De même, la CNIL a validé le principe du rassemblement des données issues des SI covid dans le SNDS lors de l'examen du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires-

ces systèmes d'information ayant en outre par construction une nature temporaire, qui n'appelle pas de dispositions codifiées dédiées. Il n'y a notamment pas lieu de restreindre l'accès aux données de contact des personnes- nom, prénom, coordonnées telles qu'adresses postale et électronique -, dès lors que ces données n'ont pas vocation à figurer dans le SNDS, celui-ci reposant sur la réutilisation de données pseudonymisées. En outre, il ne nous semble pas opportun de prévoir que les données recueillies dans les SI covid ne peuvent être conservées au-delà de trois mois que dans les conditions prévues par les dispositions du code de la santé publique relatives au SNDS, car la possibilité de prolonger la durée de conservation des données est prévue de manière plus large, dans le décret du 12 mai 2020, pour les données traitées à fins de surveillance épidémiologique ou de recherche sur le virus hors SNDS.

collectivement ou individuellement aux personnes concernées, devront être mises à jour sans qu'il soit besoin de le préciser dans le présent projet de loi. De même, il est prévu que la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en tant que responsable du traitement du SNDS et dans le cadre de l'élargissement de ce système, informe collectivement et individuellement l'ensemble des personnes dont les données sont concernées. Il me faut préciser enfin que la mise en oeuvre d'une information individuelle, pour les personnes dont les données sont d'ores et déjà enregistrées dans les SI covid, se heurte à une difficulté technique majeure application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, les données nominatives collectées dans les SI covid et qui permettraient de contacter individuellement les personnes concernées sont effacées dans les trois mois à compter de leur collecte. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons revenir à la rédaction initiale de l'article 5. est à Mme Esther Benbassa. Le présent article autorise l'intégration des données recueillies dans les systèmes d'information Sidep et Contact Covid au système national des données de santé.

1461-1 du code de la santé publique, contre trois mois pour les systèmes Sidep et Contact Covid.

relève d'ailleurs des risques pour les droits fondamentaux des citoyens quant à l'utilisation qui sera faite des données recueillies dans le cadre du pass sanitaire. Nous déplorons que le texte ne prévoie actuellement aucune garantie concernant la conservation de ces données personnelles de santé. Celles-ci sont beaucoup trop sensibles pour que l'on se prive de se pencher sur la question de l'encadrement de leur utilisation et de leur conservation.

à la manière dont ces données seront ainsi intégrées. À l'issue des travaux de la commission des lois, il faut reconnaître de nettes améliorations rédactionnelles, qui répondent à une partie des interrogations

La loi du 11 mars 2020 a autorisé, dans le respect du RGPD et sous certaines conditions, la mise en oeuvre des systèmes Sidep et Contact Covid. La durée de conservation des données de santé collectées par le biais de ces deux systèmes de traitement était initialement de trois mois ; elle a été prolongée jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer la surveillance épidémiologique et de permettre la recherche sur le virus. Or l'intégration de ces données dans le SNDS aurait pour conséquence de porter leur durée de conservation jusqu'à vingt ans. Bien que l'objectif recherché soit louable au regard de la finalité du SNDS- je pense notamment à la recherche -, cette nouvelle durée de conservation n'est pas anodine et soulève des interrogations quant au respect des exigences du RGPD. le législateur a fait le choix de ne pas exiger de consentement pour verser les données personnelles de santé dans les traitements Sidep et Contact Covid, il ne peut en être de même pour transférer ces données dans un traitement général rassemblant les principales bases de données de santé publique.

Le Gouvernement ne sera pas surpris que la commission souhaite conserver sa rédaction ; elle y est aussi attachée que le Gouvernement à la sienne. À ce stade, c'est le Sénat qui s'exprime et je vous propose, mes chers collègues, de rejeter l'amendement n° 55 du Gouvernement.

ne permet pas d'identifier la personne à laquelle se rattachent les données ; en revanche, il permet de faire la jonction entre des données recueillies par des systèmes d'information différents concernant la même personne. Cette jonction est intéressante

de dérogation ou d'adaptation concernant un certain nombre de procédures administratives ou juridictionnelles. Notre rapporteur, suivi par la commission, a préconisé de mettre fin

les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle. Dès lors, il s'agit d'un dispositif propre à la crise que nous traversons. Il est évidemment essentiel de donner aux juridictions les moyens de continuer à fonctionner dans le respect des règles sanitaires- nous nous rejoignons tous sur ce point. Par ailleurs, il s'agit d'une simple faculté faculté laissée à l'appréciation des juges ; ces derniers peuvent toujours décider que l'audience ou l'audition se tiendra en présentiel. Dans ce contexte particulier, il n'apparaît donc pas nécessaire de recueillir l'avis des parties.

La loi 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu notamment des adaptations au nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée et des contrats de mission, ainsi qu'au qu'au calcul du délai de carence entre chacun de ces contrats. Le présent amendement a pour objet de supprimer la prorogation envisagée de ces mesures. Nous sommes là totalement hors du principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

à des CDD de moins d'un mois a explosé de 250 %. La loi du 17 juin 2020 a ouvert la possibilité de déroger à la réglementation qui encadre justement le renouvellement

Les parlementaires du groupe Les Républicains sont d'accord avec le Gouvernement concernant cette disposition puisqu'en commission seule la date limite d'application des dérogations a été avancée au 15 septembre 2021. La possibilité pour un accord d'entreprise de modifier le nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée et des contrats de durée de travail temporaire n'a pas été modifiée et les salariés déjà lourdement affectés par la crise sanitaire vont connaître une précarité précarité renforcée. Nous refusons que l'on se serve du prétexte sanitaire pour s'attaquer au code du travail, qui garantit la protection des salariés. Quel

d'autoriser les partenaires sociaux à fixer le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire au niveau de l'entreprise plutôt qu'au niveau de la branche, comme le prévoient les textes de droit commun. Les dispositions permettent aussi d'ajuster, également par accord d'entreprise, la période de carence. Ces dispositions sont nécessaires pour faciliter la reprise économique et favoriser le maintien de l'emploi. Elles permettent de prolonger les relations de travail qui n'ont pas pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension de ces contrats, au titre, notamment, de l'activité partielle. L'objectif est ainsi de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la reprise de l'activité, notamment après les périodes d'activité partielle, surtout dans un contexte où les entreprises devront être en mesure de pourvoir rapidement à des besoins en main-d'oeuvre nouveaux pour répondre aux commandes et nécessités du marché. Nous le constatons, un certain nombre de secteurs sont d'ores et déjà confrontés à ces difficultés. Les partenaires sociaux doivent pouvoir ajuster, pour leur entreprise, au plus proche de leurs besoins, les règles relatives aux contrats courts. Ces dispositions s'inscrivent donc dans le cadre d'un dialogue social

de vote. C'est une erreur stratégique de la part du Gouvernement de croire que l'on peut consolider les emplois et les compétences en développant la capacité d'accroître la précarité.

Vous avez créé une économie vulnérable, instable, où la plupart des emplois sont tellement précarisés qu'ils n'attirent plus

de repos par les salariés à une date fixée par l'employeur. Ainsi, alors que ce dispositif devait prendre fin le 30 juin 2021, le texte tend à le prolonger jusqu'au 15 septembre 2021. Les présentes dispositions affaiblissent, une fois de plus, le code du travail et sont particulièrement attentatoires aux droits des salariés. Or, compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, ces mesures ne sont nullement justifiées. Disons-le clairement, nous traitons ici des mesures permettant une sortie de crise de la covid-19 dans des conditions optimales, respectueuses de l'ordre public sanitaire, afin que l'activité sociale et économique du pays reprenne progressivement jusqu'à la normale. Je vous incite, mes chers collègues, à être collectivement vigilants

peut imposer aux salariés. La commission des lois est revenue sur cette augmentation, mais elle a maintenu la possibilité pour les employeurs d'imposer six jours de congé jusqu'à la fin de l'année. Entre le Gouvernement et Les Républicains, c'est le jeu des sept différences ; mais, en l'espèce, les différences sont des nuances. Non seulement la possibilité d'imposer des jours de congé est une remise en cause du droit fondamental au repos et au respect de la vie familiale, mais surtout l'argument utilisé pour maintenir ce dispositif est fallacieux : faire croire que la reprise de l'activité économique pourrait être remise en question par les salariés qui partent en congés le 15 août est une ineptie Il est évident que les salariés de l'hôtellerie, de la restauration et des nombreux métiers de la période estivale veulent retourner au travail plutôt que de toucher 84 % de leurs revenus nets en étant au chômage partiel. Si vous demandez à ces personnes de travailler pour un salaire complet, dans ces secteurs ! Notre crainte est de voir ces mesures exceptionnelles perdurer après la crise sanitaire, sur la base d'arguments pseudo-économiques. La reprise de l'activité économique ne saurait justifier le maintien de dispositifs exceptionnels dérogeant droit du travail. Tel est le sens de notre amendement de suppression des alinéas 40 et 42. Quel La commission a essayé de trouver un bon équilibre entre le dialogue social, les exigences de la vie familiale, la possibilité de prendre des congés et l'intérêt de l'entreprise, qui est aussi- rappelons-le -l'intérêt de ses salariés. Par conséquent nous avons émis un avis défavorable

Le calendrier d'une sortie de crise, à l'époque, était évidemment difficile à anticiper. Afin de trouver pleinement leur utilité, les mesures sur les congés et jours de repos prises par ordonnance du 25 mars 2020 doivent donc être reconduites, compte tenu de la prolongation de la crise sanitaire, pour accompagner les entreprises jusqu'à la sortie de cette crise. Le Gouvernement souhaite doter les entreprises des outils nécessaires dans cette période de reprise qui s'ouvre et que nous appelons tous de nos voeux. Il s'agit donc de permettre à l'employeur de mieux gérer les périodes de congé au sein de ses équipes et d'éviter que celles-ci n'interviennent

des mesures de l'ordonnance de mars 2020 précitée, nous proposons de porter le plafond de jours de congé pouvant être imposés dans des conditions dérogatoires à huit jours, contre six précédemment. Il s'agit ainsi de permettre à l'employeur de mieux gérer les périodes de congé au sein de ses équipes et d'éviter que celles-ci interviennent toutes au moment des pics de reprise. Beaucoup d'employeurs ont utilisé cette possibilité, comme je l'ai souligné en évoquant les accords de branche et les accords d'entreprise qui traitent d'ores et déjà de ce sujet. Pour que la prolongation soit pleinement utile, il est nécessaire d'augmenter légèrement le nombre de jours de congé pouvant être imposés par l'employeur. En effet, les compteurs ne repartent pas à zéro avec la période qui s'ouvre, et certaines entreprises ont déjà largement utilisé les possibilités qui leur étaient offertes. Je me permets de rappeler, une fois encore, que tout cela doit se faire, évidemment, dans le cadre du dialogue social et avec l'accord des partenaires sociaux.

secrétaire d'État. L'objet du présent amendement est de repousser d'un mois la date limite de réalisation des coupes Aggir-Pathos pour la prise en compte de la détermination des financements des tout en restant compatible avec le calendrier d'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En effet, les financements du forfait soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées

ans. Les établissements qui doivent réaliser ces évaluations en 2021 doivent les faire avant le 30 juin afin qu'elles soient prises en compte dans le calcul des financements dès 2022. cette prise en compte n'interviendra qu'en 2023. Or les médecins coordinateurs des Ehpad, qui préparent ces évaluations et les médecins des agences régionales de santé, qui les contrôlent,

Si le vote de cet amendement peut nous donner un peu d'espoir que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les personnes âgées sera remis à niveau pour l'année 2022, je crois qu'il faut l'adopter. Telle est en tout cas la position de la commission des lois.

Puissat. Cet amendement porte sur l'obligation pour l'employeur de réaliser tous les six ans un entretien professionnel comportant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

du mien, qui le satisfait partiellement. Déjà repoussée par deux fois en raison de la crise sanitaire, qui a rendu difficile la réalisation des entretiens professionnels, l'échéance de l'obligation de l'entretien professionnel de bilan à six ans est une garantie pour les salariés. Il est important que cette échéance reste fixée au 30 juin.

les grandes entreprises ont, en moyenne, versé 140 % de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Cette générosité repose largement sur les aides publiques que les entreprises continuent de toucher le chômage partiel, les plans d'urgence ou de relance. Ainsi l'entreprise Sanofi prévoit-elle de verser 4,8 milliards d'euros de dividendes après avoir annoncé un plan de licenciement de 2 700 emplois en Europe, dont 364 postes en recherche et développement en France. Alors que le Gouvernement veut durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs au nom du déficit public, 200 milliards d'euros d'aides publiques partent en fumée dans des entreprises fantômes et dans les poches des actionnaires. Les entreprises doivent s'engager à ne pas licencier pour obtenir les aides publiques. À défaut, elles

Il y a un an, au printemps 2020, la ministre du travail de l'époque, Muriel Pénicaud, avait indiqué que l'État français demanderait aux entreprises dont il est actionnaire de ne pas verser de dividendes par solidarité. Pourtant, les grandes entreprises françaises devraient verser 52 milliards d'euros de dividendes en 2021, soit une progression de 42 % par rapport à l'an dernier.

Ces deux entreprises ont pourtant bénéficié de la baisse des impôts de production, du chômage partiel, du plan de relance aérien et des achats d'obligations de la Banque centrale européenne. centrale européenne. Plusieurs groupes dont l'État est actionnaire ont engagé d'importants plans de suppressions d'emplois alors même qu'ils figurent parmi les plus aidés par la puissance publique

la fin de l'état d'urgence sanitaire, il nous semble prématuré que des enfants et des jeunes, dont chacun sait qu'ils sont plus vulnérables que d'autres, sortent du dispositif d'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance. Nous proposons donc de proroger jusqu'à septembre 2021 le dispositif qui interdit la sortie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance pour ne pas les priver de l'accompagnement dont ils bénéficient. Un certain nombre d'entre eux sont dans des parcours d'insertion professionnelle-

de leur majorité. C'est le même mécanisme de compensation que le Gouvernement adoptera dans une loi de finances à venir pour compenser, une fois de plus,

que le Gouvernement a fait en sorte que cette mesure soit adoptée et qu'elle soit financée à hauteur de 50 millions d'euros ! En outre, je me suis engagé devant vous à ce qu'elle soit compensée lors de discussions budgétaires à venir. Vous me demandez

! Par conséquent, je considère que la garantie qui est apportée est la plus élevée possible, à ce stade de la discussion. Il appartiendra au Gouvernement comme au Parlement de veiller à ce que la loi de finances se conforme réellement à ce qui est écrit dans cet amendement. Sous cette réserve, et avec la confirmation que M. le secrétaire d'État voudra bien nous donner qu'il s'agit là d'un engagement politique du Gouvernement, j'émettrai un avis

Mme Éliane Assassi. Dans un rapport parlementaire sur le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire, remis le 14 décembre dernier à l'Assemblée nationale, les députés s'inquiétaient « de la multiplication des habilitations sollicitées par le Gouvernement pour légiférer par ordonnances relevaient que pas moins de 77 ordonnances avaient été publiées depuis le début de la crise sanitaire. Au total, ce sont 95 ordonnances qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 7 vise à en proroger une grande partie. Si l'on ajoute les éventuels règlements locaux, les Français ont été confrontés depuis dix mois à un enchevêtrement de textes et à des situations dont il était parfois difficile de déterminer le régime juridique applicable. Celui-ci peut, en effet, dépendre du jour, de la période et de l'endroit où l'on se trouve, en métropole ou dans les outre-mer, dans les Alpes-Maritimes ou dans le Gard. Ces deux effets cumulatifs, temporel et géographique, rendent difficilement intelligible le régime applicable, selon Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit public à l'université Jean-Moulin Lyon 3 et spécialiste des états d'exception. Elle explique, y a « une compulsivité normative des pouvoirs publics, une tendance à administrer par la norme », et elle poursuit, « on a l'impression que comme ils n'arrivent pas à gérer la situation, ils compensent par le normatif. Mais de ce fait, on se retrouve avec une sorte de monstre normatif, et sans investissement dans l'implémentation, la mise en oeuvre Il résulte de cette accumulation de textes normatifs et d'ordonnances une instabilité et un manque de bon sens. C'est pourquoi nous ne pouvons accepter une énième prorogation de ces ordonnances qui, dans l'ensemble, même si quelques bonnes mesures ont été reconduites- je tiens à le redire -, restreignent les droits des Français. Quel est l'avis de la commission ? La commission a déjà modifié cet article qui ne contient plus qu'une seule habilitation en matière d'activité partielle et qui permet un accompagnement progressif de la sortie de crise. Le reste des dispositions

La branche des bureaux d'études, par exemple, a indiqué que les consultants d'une même équipe pouvaient avoir des spécialités différentes. Il est donc nécessaire de pouvoir adapter le taux d'activité de ces consultants aux besoins de l'entreprise, lors de la reprise d'activité. Cette habilitation à agir par ordonnances est

vise à rétablir l'habilitation permettant au Gouvernement de prolonger par ordonnance l'année blanche des intermittents du spectacle.

mois d'août 2021. Cette prolongation est actuellement prévue jusqu'au 31 décembre 2021, mais pourrait être réévaluée si de nouvelles restrictions devaient être imposées au secteur culturel. L'habilitation à légiférer par ordonnances est donc essentielle, car elle nous permettra d'adapter la durée de la prolongation, si la situation des intermittents se révèle très difficile à la fin de l'été prochain, du fait de nouvelles restrictions. Nous souhaitons également

crise que les autres intermittents. Par conséquent, cette habilitation contribuera à accompagner la reprise de l'activité dans le secteur culturel, en prorogeant les mesures spécifiques en matière d'indemnisation des intermittents du spectacle. Dans cette perspective, la prolongation de l'année blanche est essentielle, tout comme l'adaptation des critères d'accès au régime d'assurance chômage des intermittents, prévue pour les jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail pendant la crise sanitaire.

prendra fin le 1 juin 2021, concomitamment à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin de protéger les locataires dans le contexte de crise économique et sociale actuel, le présent

l'amendement n° 18. Depuis le début de la crise sanitaire du covid-19, à l'origine de la crise sociale et économique que le pays connaît actuellement, crise qui a fortement accentué les difficultés que rencontrent les populations les plus fragilisées, les risques d'impayés se se sont renforcés ; ils concernent aussi bien les loyers que les factures d'électricité, de gaz et de chauffage. C'est pourquoi, à rebours de la démarche de la commission des lois, nous avons déposé le présent amendement, qui vise à protéger les ménages jusqu'à la fin de la prochaine trêve, le 31 mars 2022. le 31 mars 2022. Nous estimons en effet que, dans un contexte sanitaire et social toujours très difficile, il est primordial de sécuriser les situations des familles les plus exposées, alors que le Gouvernement prévoit de lever progressivement les mécanismes de soutien économique. À cette fin, cet amendement tend à prolonger la trêve hivernale des loyers et à interdire les coupures d'électricité, de gaz et de chauffage durant la période qui sépare la promulgation du présent texte et le début de la prochaine période de trêve hivernale.

Nous ne voulons pas qu'à la précarité accrue que subissent de trop nombreux salariés du fait des différents confinements et de la baisse d'activité s'ajoute l'angoisse d'une expulsion et d'une mise à la rue aux conséquences trop lourdes pour les familles.

Nous demandons donc par cet amendement la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 octobre prochain, afin de répondre à l'urgence sociale. Les

sont interdites. En effet, au regard de la situation sociale qui découle de la crise sanitaire et économique actuelle, et considérant que la trêve légale est en vigueur du 1 novembre au 31 mars, nous proposons de sécuriser les ménages durant la période qui sépare la promulgation du présent texte et la et la fin de la prochaine période de trêve. Dans un contexte sanitaire qui demeure difficile, et alors que les mécanismes de soutien économique qui devraient en compenser les effets vont commencer à être progressivement levés, il s'agit d'apporter un élément de sécurité et de visibilité aux familles les plus en difficulté.

nous proposons d'interdire les coupures de gaz et d'électricité pour l'ensemble de l'année 2021 et les trois premiers mois de l'année 2022, en inscrivant directement ce principe dans l'article 7 de ce projet de loi. Il s'agit ainsi de le rendre immédiatement applicable. Nous souhaitons que nos concitoyens les plus précarisés soient mis sous protection publique et que leur accès aux produits de première nécessité que sont l'eau et l'énergie soit garanti.

La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, considérant que le retour à la normale doit s'accompagner de l'application du droit commun en matière de trêve hivernale : celle-ci, comme son nom l'indique, est faite pour éviter de mettre des gens à la rue l'hiver et non l'été. La question de principe qui nous est posée est la suivante : qui doit prendre en charge financièrement les difficultés sociales de nos compatriotes

Je pense par exemple aux retraités de l'agriculture, de l'artisanat ou du petit commerce qui n'ont pas cotisé pendant leur vie active pour toucher des retraites importantes ; ils se retrouvent avec une petite pension et ne vivront réellement au niveau du SMIC

: il vaut bien mieux s'en remettre à des dispositifs de solidarité que d'imputer la charge de cette solidarité à des personnes qui mériteraient elles-mêmes d'en être bénéficiaires. C'est pourquoi notre commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

l'hypothèse d'une hausse à venir ne peut pas être totalement écartée à ce jour. Nous restons donc évidemment vigilants face à cette perspective. C'est pourquoi la rédaction du présent alinéa 7 est prudente permettre d'ores et déjà la prise de mesures rapides et protectrices en faveur des ménages qui seraient financièrement précarisés en cas de matérialisation d'une telle éventualité dans la période qui sépare la fin de l'état d'urgence du 31 octobre 2021, date du début de la prochaine trêve hivernale. Par conséquent, nous sommes défavorables à ces trois amendements. Pour les mêmes raisons, nous sommes également défavorables aux amendements n 45 et 97. Là aussi, la rédaction prudente de cet alinéa permet de

n'est pas exact : elle ferait peser la charge sur la collectivité publique. S'agissant de personnes éprouvant des difficultés sociales, une telle mesure n'est pas totalement illégitime, même si je reste persuadée

ce n'est pas grave ! La crise que notre pays subit depuis plus d'un an n'est pas simplement une crise sanitaire. Travailler à la sortie de la crise sanitaire, c'est bien évidemment aussi décider de mesures d'accompagnement social,

Le dispositif proposé se veut une réponse aux conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons, afin de permettre aux entreprises les plus touchées d'être accompagnées au mieux, de manière simple et rapide, et de pouvoir poursuivre leur activité avec un échéancier de dette plus soutenable. Cette procédure de traitement de sortie de crise est destinée aux petites entreprises qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique. Ainsi, nous entendons leur permettre de rebondir, grâce à une restructuration de leur dette. serait ouverte sur demande aux entreprises qui seraient en état de cessation des paiements, mais en mesure de présenter un projet de plan de continuation de l'activité. Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise donc à soutenir ces entreprises en leur permettant de continuer leur activité. Il est important de leur donner une vision plus sereine de leur avenir. Il faut faire pareil

telle prolongation d'un dispositif expérimental doit être replacée dans un contexte plus large, notamment celui de la lutte contre la précarité des travailleurs titulaires de contrats courts. Dans tous les cas, cela doit faire préalablement l'objet, me semble-t-il, de discussions avec les partenaires sociaux.

Cette disposition vise à sécuriser juridiquement une option que les maires pourraient vouloir mettre en place en mobilisant des espaces extérieurs couverts nombre d'opérations électorales ont lieu dans des écoles. C'est une mesure de simplification qui ne doit pas coûter plus cher que l'organisation classique du bureau de vote à l'intérieur. La disposition que vous avez introduite à cet alinéa, monsieur le rapporteur, constitue en revanche une charge nouvelle pour l'État,

Monsieur le secrétaire d'État, cet avis sera défavorable, mais je veux vous rassurer sur l'application correcte des règles d'irrecevabilité financière. En effet, l'article L. 70 du code électoral dispose déjà ceci : « Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État. » Si nous avons introduit cette disposition à cet article, ce n'était pas pour créer une charge nouvelle, mais simplement pour préciser que la charge nouvelle que vous créez se voit bien appliquer l'article L. 70 du code électoral.

partage la volonté de tout mettre en oeuvre pour faciliter le vote par procuration aux prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 et souscrit donc à la reconduction de ce dispositif. Toutefois, afin de ne pas solliciter déraisonnablement les officiers et agents de police judiciaire, le présent amendement a pour objet de préciser que l'électeur accompagne sa demande d'établissement d'une procuration à domicile d'une attestation sur l'honneur de son incapacité à se déplacer en brigade ou en commissariat en raison d'une maladie, dont la covid-19, ou d'une infirmité graves. Il s'agit de faire confiance à l'électeur, qui est tout à fait apte à juger de son impossibilité physique à se rendre en commissariat ou en brigade, tout en le responsabilisant au moyen de l'attestation sur l'honneur. Quel est l'avis de

la télévision ou de la radio, assurera donc une couverture large, aussi bien au niveau national, sur les chaînes linéaires et numériques, qu'au niveau local. Outre le traitement quotidien de la campagne électorale dans les tranches d'information des antennes nationales et locales, ainsi que les spots d'information sur les compétences des régions et des départements, des débats diffusés à la télévision et à la radio seront notamment organisés entre les candidats aux élections régionales avant chacun des deux tours de ces élections. Un traitement spécifique des élections départementales sera également mis en place, adapté à la spécificité de ce scrutin, ce qui n'était pas prévu dans le texte initial. Cet amendement vise donc à rééquilibrer la couverture audiovisuelle des deux scrutins et à préciser les obligations qui relèvent du service public et s'exerceront sans préjudice de la couverture médiatique prévue par les opérateurs privés ; rappelons qu'il y avait aussi eu des débats sur le rapport entre opérateurs publics et privés.

cas pour 100 000 habitants au 16 mai dernier ; la dynamique épidémiologique reste en forte hausse, enregistrant une augmentation de plus de 30 % en une semaine ; les hospitalisations et admissions en réanimation sont à un niveau élevé, avec, sauf erreur

l'annulation de l'élection prévue dans cette collectivité au mois de juin 2021, si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue, et son report au plus tard au mois d'octobre 2021. La décision d'annulation de l'élection serait prise par un décret publié, au plus tard le 12 juin 2021, après avis circonstancié du comité de scientifiques, institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, sur l'état de l'épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires liés à la tenue du scrutin, et après information de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avis du comité sera, bien évidemment, rendu public.

Notre rapporteur a fait un travail d'orfèvre pour essayer de rendre le

de l'ouverture des urnes, que le vote électronique débute dans deux jours et que les électeurs ont reçu leurs identifiants aujourd'hui, de préciser les pays où nous avons la certitude que les élections ne pourront pas se tenir.

c'est de préciser là où, de manière certaine, il n'est pas raisonnable de tenir des élections. Quel est l'avis de la commission ?

consistant à faire appel aux délégués consulaires élus voilà maintenant sept ans, qui seront les grands électeurs et n'auront d'ailleurs pas d'autre fonction

l'avis du Gouvernement ?

C'est l'autorité administrative qui prendra la décision, en constatant l'impossibilité d'organiser les élections dans un territoire donné. Elle le fera sous le contrôle du juge administratif.

des titulaires de pensions de retraite françaises vivent à l'étranger. Ils se rendent en France, par exemple pour leurs vacances, et tombent malades.

maladie. Le Gouvernement a alors eu la bonne idée de prendre une instruction assouplissant l'application de ce texte législatif. Mais cette instruction a été attaquée devant la juridiction administrative, qui n'a pas manqué de relever qu'elle était illégale et l'a donc annulée. Dès lors, les souplesses que le Gouvernement lui-même avait décidé d'appliquer dans la mise en oeuvre du texte législatif qu'il avait fait voter ont disparu. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement est-il prêt à à revenir, par une disposition législative, sur l'excès de rigueur de la loi, en prenant en compte l'instruction qu'il avait lui-même élaborée et en la « transposant

peu réaliste au regard des actions à mettre en place à la suite de ce jugement, je me permets de noter sur le fond que, selon le Conseil d'État, la condition d'une durée minimale de cotisation à un régime français permettant d'ouvrir le droit à la prise en charge des frais de santé est essentielle pour concilier l'exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics et le droit à la protection de santé et, ainsi, assurer la pérennité de notre système d'assurance sociale. Ce jugement sera sans effet sur les personnes pour lesquelles la France reste exclusivement compétente en matière de soins de santé dans le cadre des règlements européens et des conventions bilatérales de sécurité sociale. Cela représente plus de 780 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger. Pour les pensionnés ne pouvant rester affiliés à la protection universelle maladie, l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger constitue une alternative, permettant la couverture des frais de santé en cas de séjour temporaire en France. En outre, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle que, au regard de la gravité de la pandémie actuelle, plusieurs dispositifs dérogatoires de prise en charge des frais de santé ont été adoptés. Les Français vivant à l'étranger peuvent ainsi, dès leur retour en France, bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé sans qu'aucun délai de carence leur soit applicable, et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. De même, la vaccination contre le covid-19 est accessible en France pour toute personne résidant sur le territoire,

D'autres points ont encore fait l'objet d'améliorations lors de la discussion. Tout cela est positif ! Nous avions également, dès l'ouverture de ce débat, mis en avant les sujets qui nous paraissaient importants et sur lesquels nous n'accepterions pas de transiger. Je citerai tout d'abord la prolongation de l'état d'urgence sanitaire proposée par la commission des lois et votée par le Sénat pour une durée d'un mois et demi. Nous y sommes défavorables.

L'amélioration a été notable, aussi, concernant le rôle du Parlement. Mais quand nous avons abordé la question des droits sociaux et de la protection sociale, nous ne vous avons pas non plus convaincus. Vous n'avez accepté

ce régime d'exception à peine voilé. de loi de sortie de la crise sanitaire a été amélioré par le Sénat et il nous rappelle que cette épidémie mondiale, que personne n'a vue venir,

ne veulent plus être angoissés par la perspective d'un quatrième confinement. Les salariés des Ehpad, des hôpitaux et du maintien à domicile, qui ont fait des efforts considérables, nous demandent qu'il n'y ait plus de nouveaux clusters ni de nouveaux décès ; ils nous demandent la sécurité pour avoir la liberté de sortir et de partir en vacances. Restons vigilants

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce soir, notre groupe tient à saluer les modifications apportées par le Sénat à ce projet de loi. Celles-ci lui confèrent, nous semble-t-il, une robustesse dont le texte issu de l'Assemblée nationale était Alors que la sortie de crise se dessine, nous sommes convaincus de la cohérence des dispositions proposées par notre rapporteur : l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021, puis un régime réellement transitoire du 1 juillet au 15 septembre 2021. Nous ne voulions pas de l'entre-deux proposé par le Gouvernement, qui ajoute encore de la confusion dans l'esprit des Français déjà soumis à rude épreuve. Un grand nombre de garanties ont été apportées par notre assemblée quant aux modalités de sortie de la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne le pass sanitaire. Elles apaiseront, nous l'espérons vivement, les inquiétudes souvent légitimes de nos concitoyens. Le travail de notre rapporteur Philippe Bas doit être salué ; il a su examiner ce texte avec toute la rigueur et le sérieux qu'exige la crise sanitaire que nous traversons, malgré des délais particulièrement contraints, imposés par le Gouvernement. Pour l'ensemble de ces raisons, une grande majorité des membres du groupe Les Républicains votera ce texte, tel qu'il a été modifié par le Sénat en première lecture.

une vraie sortie de l'état d'urgence. Reste la question du pass sanitaire. Une partie d'entre nous accepte celui-ci, parce qu'il permettra le retour à la vie,